dans les groupes d'études qui ont été promus par le Gouvernement et par Mme la ministre, MM. Villani et Petit et Mme Retailleau

de septembre dernier, M. le ministre de l'agriculture a déclaré vouloir mettre la souveraineté alimentaire au coeur des politiques agricoles européennes. Mon groupe se réjouit de cette perspective, car il a toujours été attentif

résolution ! Au-delà de la seule autonomie alimentaire de la France et de son caractère stratégique, nous sommes bien évidemment face à un enjeu d'ordre mondial. On estime à 9 milliards le nombre d'individus qu'il faudra nourrir à l'horizon de 2050. Le monde sera-t-il en capacité de produire les ressources nutritives nécessaires pour répondre à ce défi ? À la problématique de la dynamique démographique s'ajoute, on le sait, la question du changement climatique et de son impact sur potentiel agricole, notamment sur le continent africain. Les études prospectives montrent que, à technologie inchangée, des tensions pourraient émerger entre les pays, notamment sous la forme de conflits d'usage des terres et de l'eau. Aussi, la recherche doit s'engager à garantir l'autosuffisance alimentaire pour notre pays et à tous les États qui en auront besoin. Il faudra de nouvelles réponses techniques au défi agricole sous-jacent à la question alimentaire, un défi qui doit en outre répondre aux impératifs de développement durable. Dans le projet de loi, le rapport annexé mentionne la nécessité d'entretenir en continu la production de connaissances et énumère les enjeux essentiels : sanitaire, climatique, énergétique ou numérique. L'amendement vise à compléter cette énumération par l'enjeu alimentaire, qui, comme je viens de le dire, a grandement besoin de la science et de la recherche pour s'adapter aux évolutions du monde de demain.

actuel, est-il utile de rappeler combien la santé est prioritaire ? La recherche de solutions adaptées aux territoires et socialement acceptables doit aussi s'exercer à l'égard du défi sanitaire. Depuis le début de l'année 2020, la pandémie de covid-19 a placé la santé au coeur des priorités de la recherche, en particulier pour l'élaboration de tests et la découverte d'un vaccin. C'est également à l'échelon organisationnel que la crise a posé des défis à la recherche, par exemple avec la mise au point d'applications numériques de traçage des malades. Dans les années futures, parce qu'un virus a réussi à arrêter pendant plusieurs semaines la marche du monde, la santé devra être, encore plus qu'elle ne l'est déjà, un sujet de recherche de premier rang

». En effet, la directive européenne à laquelle il est fait référence dans cet alinéa couvre les utilisations d'animaux à des fins scientifiques et éducatives. Il convient donc, par cohérence, de rétablir cette

Conformément aux recommandations de la directive européenne, les « trois R » doivent s'appliquer dans l'ordre suivant : d'abord le remplacement, lorsque cela est possible, ensuite la réduction, si le remplacement n'est pas possible, enfin le raffinement, dans tous les cas où des animaux sont utilisés. Cette hiérarchisation des méthodes, qui date des origines du concept, est reprise dans l'article 4 et le considérant 11 de la directive européenne. La définition du remplacement n'a pas à inclure les termes « dès que possible ». Les méthodes de remplacement existantes dont la validité est attestée doivent être utilisées dès lors qu'elles sont susceptibles de permettre d'obtenir un résultat au moins aussi satisfaisant que l'utilisation d'animaux. Le fait de ne pouvoir engager des projets sur animaux que s'ils sont indispensables figure déjà dans la réglementation. Pour autant, cette obligation n'entre pas dans la définition d'une méthode de réduction. La mention de « protocoles validés » est également inutile, puisqu'un projet ne peut être autorisé par les autorités compétentes que si les protocoles concernant l'utilisation des animaux ont été validés par le comité local éthique en expérimentation animale.

que les méthodes de substitution aux expérimentations animales présentent des avantages en matière de recherche scientifique, d'une part, en apportant la possibilité de tester certaines molécules qui ne fonctionnaient pas sur les modèles animaux classiques, et, d'autre part, en offrant un taux de prédictibilité meilleur que ceux-ci. C'est l'argument que j'avançais tout à l'heure. Le problème majeur reste le nombre infime de nouveaux tests alternatifs validés. En effet, l'organisme européen chargé de la validation n'en valide guère plus d'un par an. Très peu de laboratoires de recherche se lancent dans le processus de validation réglementaire d'une nouvelle méthode, car c'est long- entre sept et dix ans -, très coûteux- de l'ordre de 100 000 à 200 000 euros -et sans aucune garantie d'un retour sur investissement, puisqu'il n'y a pas de brevet pour ces nouvelles nouvelles dispositions. À titre d'information, plus de 500 000 animaux ont été utilisés en France en 2018 à des fins toxicologiques ou réglementaires, soit un peu plus de 27 % du total des animaux utilisés. Cette volonté d'améliorer et d'accélérer les processus de validation des méthodes alternatives au test réglementaire est affichée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation dans sa réponse à la question écrite de l'une de nos collègues députés. Il est donc essentiel qu'un organisme national, tel que celui qui est prévu par ce texte, puisse inciter les laboratoires de recherche à demander la validation de nouveaux tests en oeuvrant à l'échelon national pour la réduction significative du coût et de la durée de cette démarche et en étant force de proposition à l'égard des instances européennes.

notamment à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Centre national de la recherche scientifique et à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. L'utilisation des animaux à des fins scientifiques concerne les secteurs de la santé, de la biologie, de l'environnement et de l'agronomie. Il paraît donc essentiel que les acteurs majeurs de la recherche publique dans ces domaines participent à la création et aux activités de ce centre.

en vue de cette création. À ce stade, sans anticiper sur le travail à venir, on peut préciser qu'il doit être adossé à la recherche publique, notamment notamment à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Centre national de la recherche scientifique et à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

que l'organisme puisse contribuer à l'amélioration de ce processus de validation.

mais ces propositions me paraissent prématurées, car elles relèvent du travail préparatoire à la création de l'institut. Il semble difficile de fixer dans la loi la façon dont vont s'organiser les différents organismes de recherche pour mettre en place ce centre de la manière la plus efficace possible. Je mets

de s'assurer que le centre national peut participer à la promotion des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Il me paraît nécessaire de le prévoir d'ores et déjà à travers un véritable organe de gouvernance ouvert, mais également de prévoir que le statut juridique soit particulièrement approprié pour l'ensemble de ses missions.

le Gouvernement entend créer un portail unique présentant l'ensemble des appels à projets, ce qui est une très bonne chose. Cet amendement a pour objet d'inclure le domaine de la santé dans le champ de ce portail. En effet, la santé dispose de plusieurs agences ou programmes nationaux, ce qui appelle à un regroupement sur un portail unique de ceux-ci et à une action de rapprochement de leurs modalités de gestion scientifiques et financières. Il en résultera un bénéfice pour les chercheurs, qui auront une vue globale et simplifiée des appels ouverts et après rapprochement des modalités de gestion également simplifiées. Il en résultera également un bénéfice pour l'efficacité de l'action publique, en évitant les doublons entre programmes et en facilitant leur articulation.

Il a été adopté au Sénat grâce au soutien de cent cinq sénateurs, toutes tendances politiques confondues, mais le Gouvernement et l'Assemblée nationale s'y sont opposés. Peu avant le confinement, j'ai adressé un courrier cosigné par cent quarante sénateurs à Mme Kyriakídou, commissaire européenne à la santé et à la politique des consommateurs, afin d'obtenir des financements pour soutenir la recherche, notamment en faveur d'un vaccin contre L'incidence de la maladie ne cesse d'augmenter : de 26 000 nouveaux cas en 2014, nous sommes passés à 67 000 en 2018 en France. La crise sanitaire déclenchée par l'épidémie que nous connaissons actuellement nous impose d'accroître en urgence les travaux de recherche sur les zoonoses et les maladies vectorielles à tiques, ainsi que les moyens qui y sont consacrés. Il existe plus de deux cents types connus de zoonoses. Elles sont un problème majeur de santé publique dans le monde entier, en raison de notre relation étroite avec les animaux dans différents contextes- l'agriculture, les animaux domestiques et notre environnement naturel. Les zoonoses représentent une forte proportion de l'ensemble des maladies infectieuses nouvellement recensées. Certaines d'entre elles, comme le nouveau coronavirus, ont le potentiel de provoquer des pandémies mondiales, dont les conséquences sanitaires, économiques et sociales sont sans précédent, comme on le voit voit aujourd'hui. L'amendement que je défends vise donc à créer un nouveau programme prioritaire de recherche sur les zoonoses et les maladies vectorielles à tiques, afin de consacrer des crédits spécifiques à la lutte contre ces maladies infectieuses en pleine expansion. expansion. Si je dépose continuellement ces amendements, c'est que je suis portée par des milliers de malades en souffrance, qui ne comprennent pas non plus que les médecins ne soient pas tous d'accord pour les prendre en charge. Mes chers collègues, je vous demande donc, comme à mon habitude, d'être solidaires de cet amendement.

Reconnaissez que ces interactions couvrent un continuum qui va de la diffusion de la culture scientifique auprès du grand public jusqu'au développement de recherches participatives, en associant des chercheurs et des non-chercheurs dans une démarche partagée. Cet amendement vise à structurer l'ensemble de ces interactions

L'alinéa 235 du rapport annexé prévoit la création d'un réseau « Science et médias », destiné à « permettre la mise en contact rapide entre journalistes et chercheurs » dans un but de diffusion de la culture scientifique. comprenons les ambitions et les objectifs de cette mesure, qui sont louables : il s'agit d'inventer des moyens pour promouvoir la méthode scientifique, de lutter contre les et les théories du complot et de mieux armer intellectuellement la population pour y faire face. Toutefois, c'est la méthode retenue qui nous pose problème.

Le principe est simple : ces centres sont des relais entre la communauté scientifique, d'une part, et les médias et la société civile, d'autre part, pour fournir des éclairages sur certains sujets. Au Royaume-Uni, ce centre ne fait pas l'unanimité. Un article paru dans en 2013 souligne que de nombreux acteurs considèrent

Mes chers collègues, ce dont la méthode scientifique a besoin dans notre société, c'est du débat et de la coopération, pas de la verticalité. Ces approches « verticales » de pédagogie forcée et de vulgarisation agressive ne fonctionnent pas avec ceux qui doutent de tout, y compris de la science. Ce n'est pas en apportant la lumière « sacrée » de la vérité de la science, depuis le haut du piédestal d'une énième institution ou d'un mandarin que nous parviendrons à ramener ces personnes dans un débat public raisonnable. C'est d'ailleurs précisément le rejet de tout ce qui provient de l'État, des élites ou des institutions qui conforte ces publics dans leurs positions. Il nous faut inventer de nouvelles formes de débats scientifiques, et le chemin sera long. Ce dernier passe par l'éducation, par la culture, par la coopération avec nos institutions, par la forme de nos institutions, par la manière dont nous faisons société. Mais il ne passe pas par un Centre de promotion de la science officielle, qui sera plutôt contre-productif. Quel est l'avis de la commission ? L'amélioration de la qualité de l'information scientifique est une condition essentielle à la préservation du lien de confiance entre les citoyens et les chercheurs.

le Sénat l'appréciera particulièrement - des ressources au sein des enseignants-chercheurs, auxquels les médias pourraient s'adresser pour nourrir le débat public, pour lutter contre le désordre informationnel et pour permettre à chacun de comprendre le monde qui l'entoure et d'y prendre part. Participer à ces réseaux pourra faire partie de ce qui permettra aux chercheurs et aux enseignants-chercheurs de progresser dans leur carrière. Je rejette complètement le qualificatif de « vertical », puisque cela sera construit avec les chercheurs et les enseignants-chercheurs et les usagers sur le terrain. J'ajoute que cette initiative ne relève en rien d'une pédagogie d'État. Mon ministère n'est pas le ministère de la propagande, c'est celui des chercheurs, c'est celui qui fait du doute méthodique et de la démarche scientifique leur boussole quotidienne. Enfin, je suis surprise que vous vous fassiez le porte-voix d'une association qui a refusé d'être auditionnée par l'Assemblée nationale au mois d'août dernier. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.

que je vous invite à lire comme je le fais tous les matins. C'est un média totalement libre, gratuit, sans aucune publicité et qui fonctionne grâce aux subventions de soixante établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Sa caractéristique, c'est que ce sont des chercheurs qui écrivent les articles, donc des chercheurs qui deviennent journalistes et qui, chaque matin, vous expliquent l'actualité de leurs recherches avec des mots très simples. Je pense que ce type d'initiative devrait être soutenu par votre ministère. Ainsi, je regrette que, pour ce média, les subventions publiques ne représentent que 10

paraissent louables en ces temps de crises multiples. La nécessité de penser la médiation scientifique paraît en effet très urgente, alors que nos sociétés sont face à des choix techniques de plus en plus nombreux et complexes. la solution de centres science et médias, proposée dans le texte de loi, n'est pour nous pas la bonne. On peut malheureusement craindre, avec le dispositif prévu par le texte, une instrumentalisation de la science, car la référence dans le texte de loi aux exemples étrangers est particulièrement malvenue,

de certains de ses donateurs. Ainsi, les experts mis en avant par cette agence avaient pour certains des conflits d'intérêts avérés. De plus, une large partie d'entre eux n'était même pas des scientifiques de profession. Citer ici cet exemple est-il une maladresse ?

en capacité d'instrumentaliser les discours et l'autorité scientifique dans l'espace public. Au contraire, les sciences doivent être plurielles, comme on l'a dit, madame la ministre. Plutôt que de créer un réseau d'experts, supposés légitimes, de laisser s'exprimer une diversité de points de vue scientifique, permettant aux citoyens de se faire une opinion éclairée, par le biais biais de journalistes d'investigation qui sont aussi des professionnels et que l'on doit reconnaître. On connaît les stratégies des grandes entreprises pour fabriquer du doute

supprimer la création des pôles universitaires d'innovation. Il s'agit d'un ajout de complexité, certainement pas d'une simplification culturelle. Le label « Pôle universitaire d'innovation » doit permettre de fluidifier sur un territoire donné les relations entre les acteurs de la recherche publique et ceux du monde économique, sans création de structure nouvelle. La commission émet donc un avis défavorable.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme mes collègues du groupe socialiste, que nous ayons réduit la période de planification à une durée raisonnable, et l'augmentation des budgets prévus par l'article 2 peut être saluée, même si elle pourrait être plus importante, nous y reviendrons tout à l'heure. Toutefois, avant d'examiner cet article dans le détail, je voulais vous faire part de mon sentiment global et de mon inquiétude. Ce dont la recherche française a besoin, c'est avant tout de financements pérennes. La part de l'ANR et son augmentation sont importantes : elles annoncent un recours sans cesse plus important au financement par le biais d'appel à projets. En soi, le financement par appel à projets présente parfois des avantages, mais il ne peut pas devenir la règle : c'est un modèle incertain, insécurisant et trop chronophage pour nos chercheurs. Pour Pour reconstruire un service public fort de la recherche française, il faut sortir nos chercheurs de la quête perpétuelle de financement, en donnant des moyens pour la recherche fondamentale, en créant davantage de postes de titulaires en veillant à l'égalité de traitement entre toutes nos universités, nos laboratoires et nos centres de recherches, où qu'ils soient situés sur le territoire. Nous avons les moyens de briller dans de nombreux domaines. Notre pays ne manque pas de femmes et d'hommes capables d'être à la pointe de la recherche, que ce soit en sciences physiques, en mathématiques, en biologie, en médecine, en philosophie, en histoire, littérature, en sociologie ou en économie. En outre, comment espérer que nos chercheurs puissent trouver des idées nouvelles pour répondre aux enjeux écologiques, économiques et sociaux auxquels nous devons faire face ? Hier soir, dans cet hémicycle, nous avons eu des échanges animés pour savoir si nous devions ou non réintroduire les néonicotinoïdes dans le secteur de la betterave. Mais nous savons tous que l'une des parties du problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment financé la recherche pour trouver des alternatives ! Et ce n'est qu'un exemple. Le prix à payer pour retrouver le chemin de l'excellence et inventer des solutions nouvelles pour construire notre avenir, c'est de leur donner du temps. Nous savons, dans notre société en perpétuelle accélération, que cela a un coût important, mais le jeu en vaut la chandelle ! Et je crains, malheureusement, que ce texte ne suffise pas à atteindre cet objectif.

je crois qu'il est important de souligner la nécessité d'accroître la trajectoire de création d'emplois, et d'emplois statutaires, c'est-à-dire stables. En réalité, vous prévoyez, madame la ministre, 5 200 emplois sous plafond supplémentaires d'ici à 2030. Vous avez raison, c'est bien créer des emplois.

Et, en sept ans, entre 2010 et 2018, le nombre d'enseignants-chercheurs a stagné, passant d'un peu plus de 50 000 à 50 700. Les effectifs d'étudiants et à l'université ont pendant ce temps-là augmenté de 14 %. Vous le voyez bien, nous sommes dans une situation où, déjà, globalement, le nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs a tellement diminué que l'accroissement que vous prévoyez ne nous remet pas à flot, sans compter que s'y ajoute toute une série de contractuels, qui développent une précarité qui ne nous paraît pas de bon augure pour faire de bons chercheurs.

en capacité de recherche ou est-ce qu'on limite la casse en continuant le déclin ? » Car c'est cela, le risque qui nous menace ! Je ne dis pas que c'est écrit d'avance, mais, ce qui est clair, c'est que sans un sursaut aujourd'hui sur les trajectoires d'emplois et sur les moyens budgétaires, il y a des risques de déclin pour notre nation, alors même que l'on a les moyens d'un sursaut. J'entends bien les problèmes budgétaires, mais j'observe que, dans certains secteurs, il n'y a pas de problème- j'ai parlé de certains avantages fiscaux ici ou là -et que dans d'autres, ce serait irréaliste, pas raisonnable. Pour ma part, je crois que ce qui serait irréaliste et pas raisonnable, ce serait de ne pas donner le coup de collier qui s'impose, en termes d'emplois et de budget, au profit de la recherche nationale.

Le financement pérenne des structures de laboratoire n'est pas contradictoire avec le modèle de l'appel à projets. C'est un choix, et Mme la ministre a rappelé les proportions.

qui va être rappelé à plusieurs reprises dans ce débat, et j'en suis désolé, mais je dois tout de même le dire, comme je l'ai dit pour la partie budgétaire, ce n'est pas au moment où l'on veut corriger le tir

? Oui ! Non, non, non, cher collègue Pierre Ouzoulias ! Est-ce que la France a fait des progrès avec le modèle mixte ? Guère plus,

Mais permettez-nous d'explorer toutes les voies de la recherche, y compris en matière

le surcoût imposé à la masse salariale des emplois, des établissements et des universités. Aujourd'hui, cela représente des montants extrêmement importants.

juin 2020, le Conseil économique, social et environnemental souligne : « [Sous] l'effet de l'augmentation mécanique du PIB en lien avec les cycles économiques de moyen terme et de l'inflation à cet horizon de dix ans, cette hausse de la dépense publique ne permettra pas d'atteindre, malgré la récession prévue en 2021, voire 2022, l'objectif de 3 % que la France s'était fixé il y a vingt ans et qui permettrait de redonner le souffle nécessaire à la recherche française. nécessaire à la recherche française. » La France s'est engagée à investir 1 % de son PIB dans la recherche publique. Selon le collectif des sociétés savantes académiques de France, dans un scénario de 1 % de croissance annuelle moyenne du PIB et de 1 % d'inflation, le PIB de 2030 atteindra 2 900 milliards d'euros Dans ce scénario réaliste, ce sont donc près de 12 milliards d'euros courants additionnels, et non 5 milliards d'euros, qu'il faudrait ajouter au budget annuel de la recherche publique à l'horizon de 2030.

rectifié . La trajectoire budgétaire du Gouvernement a tout de même le mérite de rompre avec des décennies de sous-investissement chronique dans la recherche. Ce changement de cap va enfin donner à ce secteur des marges budgétaires nouvelles et de la visibilité à moyen terme. Néanmoins, comme je le pointe également, le niveau de réinvestissement proposé sur dix ans ne permettra pas d'atteindre l'objectif de 3 % de dépenses en faveur de la recherche, dont 1 % de dépenses publiques. Avec mes collègues rapporteurs pour avis, nous avons donc fait le choix de ramener à enveloppe constante la programmation à sept ans, de permettre une montée en charge plus rapide des moyens nouveaux, en particulier au cours des deux prochaines années. Nous aurions évidemment aussi pu proposer d'augmenter le montant de l'enveloppe globale, mais nous tenions à présenter une alternative forte et crédible. Le projet des auteurs de l'amendement est généreusement ambitieux. Mais est-il crédible à l'heure où nous traversons une crise sanitaire et économique sans précédent qui exige d'abonder d'autres secteurs ? L'amendement secteurs ? L'amendement n° 59 rectifié vise à présenter la trajectoire budgétaire en euros constants. Comme l'indiquent à juste titre les auteurs, la présentation de cette programmation en euros courants ne permet pas d'intégrer les effets de l'inflation.

Je le précise, quelque 500 millions d'euros ont été consacrés exclusivement aux universités dans les précédents budgets, afin d'accompagner la montée en puissance du nombre d'étudiants. Au reste, celle-ci était prévisible depuis les années 2000

voulons augmenter de 30 % le montant des contrats doctoraux. La vie étudiante est évidemment essentielle. Le Gouvernement y consacrera 134 millions d'euros supplémentaires dans le projet de

tout de même un peu fort qu'un membre du Gouvernement aille contre les propositions budgétaires des autres ministères. Toutes les lois de programmation sont à sept ans. Et

contre le CNRS, sa bureaucratie et ses multiples laboratoires dont quelques chercheurs décidaient « quelquefois démocratiquement

Vous avez senti qu'il était nécessaire de redonner confiance à tous les chercheurs, dans toutes les institutions où ils

cet amendement est d'intégrer à la partie normative de la loi de programmation l'évolution planifiée des effectifs en équivalents temps plein travaillé, ou ETP. En effet, l'une des craintes les plus vives exprimées par le monde de la recherche est que les nouvelles voies de recrutement créées par ce texte, telles que les chaires de professeurs juniors, le contrat doctoral de droit privé ou le CDI de mission, ne viennent purement et simplement se substituer aux emplois traditionnels de la recherche.

le budget de l'État contribue très largement, par des mécanismes de financement directs ou indirects, à la recherche et au développement des médicaments arrivant sur le marché. L'État finance un système d'enseignement supérieur d'excellence qui forme les scientifiques et les chercheurs. Il

les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne, la Suède et la Grande-Bretagne ont investi plus de 870 millions d'euros dans la recherche sur les vaccins, traitements et diagnostics contre la covid-19, alors que la France a déjà investi plus de 57,25 millions d'euros à ce titre. Quant à la recherche sur les vaccins candidats, l'Union européenne a déjà contribué à hauteur de 400 millions d'euros pour le, ou Covax. De même, la France a signé des accords bilatéraux de préachat de doses de vaccins candidats, lesquels sont aujourd'hui indisponibles à la consultation du public.

L'objectif de cet amendement est d'améliorer la transparence des marchés relatifs aux médicaments, vaccins et autres produits de santé, et de veiller à ce que les informations soient publiées. L'instauration de la transparence permettra d'apprécier la fixation des prix des médicaments à l'aune des fonds publics En effet, il est anormal que le prix des médicaments ne tienne pas compte de tous les investissements publics qui ont pu être faits. La transparence ne saurait être garantie sans la mise à disposition de ces informations au public. La création d'un répertoire qui pourra être consulté par tous y pourvoira.

du PIB et qui profite en bout de chaîne aux entreprises et à l'industrie. Dans le contexte de la crise de la covid-19, une partie de la recherche publique est fortement mobilisée pour la découverte d'un vaccin.

Compte tenu de l'échelle de la pandémie, les enjeux financiers liés à la fabrication d'un vaccin sont considérables. Il règne pourtant, de manière générale, une certaine opacité sur les négociations entre l'État et les laboratoires, notamment sur la fixation du prix d'un médicament. Pour des raisons éthiques et pour contribuer à la soutenabilité financière de notre système de santé, il serait souhaitable d'introduire davantage de transparence et de mettre en valeur les bénéfices que la recherche publique garantit à ceux qui sont en charge du transfert de technologies.

nous examinons affiche l'objectif assez ambitieux de porter progressivement à 1 % du PIB la part du financement du régime public de la recherche.

de 6 milliards d'euros en 2019, et le CICE, qui a bénéficié à hauteur de 100 milliards d'euros aux entreprises, depuis 2013. De tels montants, issus de l'argent public et distribués à des acteurs dont le but principal est le profit, méritent d'être mieux encadrés.

pas à ceux du classement de Shanghai. Je m'interroge aussi sur la capacité de ce classement à mesurer la liberté d'expression et les libertés académiques que nous avons défendues en préambule. La

dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle, comme l'indique l'article L. 123-9 du code de l'éducation, instauré par la loi Faure de 1968. Depuis que le présent

» ; « Notre activité de recherche n'est bien souvent réalisée que pendant les congés universitaires » ; « La logique croissante des appels à projets rend cette activité chronophage et met à mal la liberté scientifique et pédagogique » ; « Les efforts à fournir pour espérer un poste, une promotion ou une reconnaissance deviennent démesurés » ; Les burn-out se multiplient » ; « L'espace de l'enseignement supérieur et de devient une machine à broyer l'humain ». Ce ne sont que quelques extraits, mais ils montrent clairement que, si l'on veut offrir les conditions d'indépendance et de sérénité nécessaires au service public de la recherche, il faut y mettre les moyens, y compris budgétaires. Quel

extrêmement attractifs. L'attractivité se définit dans un rapport entre le nombre de postes disponibles et le nombre de candidats. Or il y a aujourd'hui, dans le domaine de la recherche, une distorsion énorme entre le nombre de candidats et le nombre de postes ouverts, tellement importante que les concours de recrutement dans l'enseignement supérieur et au CNRS sont des concours de niveau international. En effet,

Madame la ministre, qui s'est consacré à ces sujets. Au CNRS, le nombre de candidats au concours de chargé de recherche est passé de 8 120 en 2011 à 5 445 en 2018, soit un tiers de candidats en moins. Sur la même période, le nombre de candidats ingénieurs et techniciens a baissé de 43 %.

que l'on est recruté une fois et que le second jury est un jury de confirmation, dont la décision est liée à celle du premier jury. J'aimerais en avoir la confirmation, parce que c'est un point extrêmement important dans notre discussion.

est parallèle au recrutement sur concours. Comme le souligne le Conseil économique, social et environnemental dans son analyse du projet de loi, ces contrats à durée déterminée sans concours, accordés sans passer par les emplois de chargé de chargé de recherche ou de maître ou maîtresse de conférences, seraient intercalés entre les postdoc et le recrutement statutaire, soumis à une simple évaluation, accroissant de la même durée la période d'emploi non permanent des docteurs.

Ces dérogations aux recrutements statutaires verront des statuts différents cohabitant sur les mêmes fonctions, ce qui ne favorise pas la cohésion du corps enseignant dans son ensemble. Nous souhaitons, au contraire, la stabilité, la cohérence et l'unité des parcours professionnels de l'enseignement supérieur et de la recherche,

disciplinaire, ne sont pas adaptées. Dans le souci de mieux affirmer le caractère circonscrit et complémentaire de ce dispositif, elle a tenu à abaisser le pourcentage de recrutements annuels autorisés par cette voie à 15 %. Elle a également souhaité mieux l'encadrer, afin de répondre aux inquiétudes exprimées par la communauté des chercheurs et enseignants-chercheurs.

pour entrer dans le corps des chargés de recherche au CNRS. J'ai été recruté, puis titularisé dans mon corps, au bout d'un an, par

madame la ministre,

commission ? L'objectif du dispositif est justement de supprimer l'étape de la qualification, afin d'avancer l'âge de recrutement des jeunes docteurs. En revanche, la commission a tenu à réintroduire une dimension nationale,

Robert. Cet amendement vise à garantir l'intérêt scientifique des recrutements des chaires de professeur junior par les instances d'évaluation compétentes des établissements concernés. L'amendement Guidez. Cet amendement vise à réduire l'utilisation des « chaires d'excellence ». L'article 3 instaure une nouvelle voie de recrutement pour les titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent avec la mise en place d'un système de prétitularisation conditionnelle. Ces « chaires d'excellence » permettraient à des contractuels de bénéficier en trois à six ans d'un passage rapide au grade de professeur ou directeur de recherche sans aucune des obligations statutaires imposées aux maîtres de conférences et chargés de recherche pour espérer atteindre le même objectif. s'agit d'une rupture complète avec le mode de recrutement national, qui passe principalement par concours de la fonction publique. Il faut noter que ces embauches, prélevées sur le même budget que les postes de professeurs des universités et directeurs de recherche, diminuent les possibilités d'évolution vers ces grades pour les maîtres de conférences et chargés de recherche. Il est donc indispensable de faire de cette voie de recrutement une exception. C'est pourquoi cet amendement tend à réduire le pourcentage maximal de recrutements autorisés chaque année dans le corps concerné de 25 % à 15 %.

Robert. L'article 3 prévoit une nouvelle voie de titularisation dans un corps de directeur de recherche. Cette titularisation est subordonnée à un engagement de servir sans que la durée de celui-ci ne soit précisée. Certes, l'article prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions de l'engagement à servir. Il est cependant souhaitable que ces conditions soient fixées dans le respect d'un cadre défini par le Parlement lui-même. S'il est important que la titularisation soit assortie d'un véritable engagement, la mobilité est également importante. L'objet de cet amendement est donc de prévoir une durée de six ans pour cet engagement de servir.

Par cet amendement, nous voulons que la commission qui décide la titularisation des chaires juniors soit la même que la celle qui organise le recrutement des maîtres de conférences. Il est important d'harmoniser le processus de recrutement. À cet égard, il est logique que, au sein d'une même université, ce soient les mêmes personnes qui se chargent de l'ensemble des recrutements, de manière à garantir une cohérence dans la politique de recrutement à l'université et une égalité de traitement entre les candidats aux différents postes. La création de ce nouveau type de contrat, directement inspiré du modèle anglo-saxon des, suscite suscite de nombreuses inquiétudes, que je partage. Au demeurant, il n'existe aucune garantie que ce dispositif renforce l'attractivité de la France pour les jeunes chercheurs, ni que ce nouveau statut de contractuel sera une sera une vraie chance pour celles et ceux qui en bénéficieront. Il risque de s'accompagner d'une augmentation du recours aux postes de vacataires pour assurer des missions d'enseignement, alors que ceux-ci sont déjà trop nombreux à être confrontés à des situations précaires. Ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui pour renforcer l'attractivité de la recherche dans les universités françaises, ce sont des créations de postes d'enseignants-chercheurs titulaires et une amélioration de la rémunération en début de carrière.

Par ailleurs, les membres du CNU n'ont pas nécessairement le meilleur profil pour faire partie de la commission : ils sont habitués à qualifier des candidats d'environ 34 ans, sur la base de publications scientifiques, alors que, dans le cas des chaires de professeur junior, il s'agira

titularisation ! Mon amendement a pour objet de supprimer du texte l'obligation de subordination à un engagement de servir pour la titularisation des chaires de professeur junior dans le corps des professeurs d'université. L'engagement de servir est une obligation réglementaire qui concerne, sauf exception, des corps classés dans la catégorie A et constitue la contrepartie d'un investissement consenti par l'administration pour leur formation. Cet engagement de servir et de rester au service de l'État est une contrepartie de la prise en charge par l'État des frais de formation et de traitements versés pendant cette formation. Ce n'est pas le cas pour les chaires de professeur junior, qui sont rémunérées pour un emploi.

Il est cependant souhaitable que ces conditions soient fixées dans le respect d'un cadre défini par le Parlement, notamment en imposant une durée de cet engagement. Il est important que la titularisation soit assortie d'un véritable engagement. L'objet cet amendement est donc de prévoir une durée de six ans pour cet engagement de servir,

de directeurs de recherche dans le grade de professeur justifie une durée de service relativement plus longue que ce que l'on a l'habitude de voir, avec parfois des demandes rapides d'exeat ou de mutation qui peuvent porter atteinte à la pérennité d'un projet de recherche.

Le Conseil d'État fixera les modalités d'application de la création des chaires de professeur junior. L'objet de cet amendement est de préciser que le décret déterminera les modalités de l'appréciation de l'habilitation à diriger des recherches des personnes concernées, par parallélisme avec les cursus de recrutement classiques, les candidats à la titularisation dans le corps des professeurs des universités devant être titulaires de cette habilitation. de cette habilitation. Madame la ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance, afin de poursuivre l'examen de ce texte. Dans la mesure où nous ne reprenons nos travaux demain qu'à dix heures et demie, nous pourrions poursuivre nos débats de ce soir jusqu'à une

Madame Guidez, la commission a déjà abaissé à 15 % le taux de recrutements annuels autorisés. Elle l'a, en revanche, maintenu à 25 % pour les corps aux effectifs très réduits, comprenant moins de cinq personnes. En effet, l'abaisser à 15 % reviendrait dans ce cas à rendre le dispositif inopérant

Sans revenir sur les apports de la commission, l'amendement n° 220 tend à préciser et à compléter utilement l'article 3, en alignant la procédure de titularisation des enseignants-chercheurs sur celle du droit commun, en précisant qu'elle relève d'un décret du Président de la République, en clarifiant la rédaction relative au taux limite de recrutement dans les corps aux faibles effectifs en enrichissant les modalités du bilan présenté par le chef d'établissement en prévoyant des données relatives à la proportion de femmes et d'hommes recrutés sur des chaires de professeur junior. Pour ces raisons,

L'amendement n° 219 du Gouvernement vise à revenir sur une précision rédactionnelle adoptée en commission, qui, à la réflexion, limite le champ des activités prises en compte pour la phase de titularisation des bénéficiaires d'une chaire de professeur junior : j'émets un avis favorable. l'amendement n° 52 rectifié, l'idée de fixer une durée d'engagement est intéressante. En effet, l'objectif n'est pas que la personne, une fois titularisée, reparte aussitôt à l'étranger. On attend d'elle un minimum d'investissement dans son corps de recrutement. Cet engagement à servir est d'autant plus important qu'une dotation publique de 200 000 euros est prévue pour chaque chaire créée. La

rectifié de M. Piednoir, qui tend à clarifier la rédaction de la condition d'obtention de l'habilitation à diriger des recherches introduite par la commission pour la titularisation dans le corps de professeur des universités.

la politique d'emploi peut être débattue en conseil académique ou en conseil scientifique, mais ces instances n'émettent que des avis simples ; ce sont les chefs d'établissement qui prennent leurs responsabilités.

68 rectifié. L'alinéa 22 prévoit le renouvellement du contrat sans en préciser la procédure. Cet amendement vise donc à indiquer que le conseil académique et le conseil d'administration, réunis en formation restreinte, se prononcent sur le renouvellement.

La séance est reprise.

nous proposons la suppression de l'article